les juifs, avec l'empereur Napoléon I ; les catholiques, en 1905, quand la République n'hésita pas à user de mesures violentes- la déportation de moines, par exemple -pour imposer à tous

Résultat, toutes les religions dont les relations avec l'État sont parfaitement apaisées et harmonisées se trouvent injustement visées par votre texte globaliste, devenu punition collective. Les croyants sont des parias et les cultes deviennent suspects.

L'esprit de nos lois est ainsi pétri de notre héritage civilisationnel, culturel, esthétique, intellectuel et religieux. Il suffit, pour s'en convaincre, de lever les yeux, sinon vers le ciel, du moins vers tout ce qui nous entoure, ici, mes chers collègues. pilier de notre République, légifère sous le regard bienveillant du roi Saint Louis ; le plafond de la salle des conférences, un véritable livre d'histoire de France, nous renvoie vers sainte Clotilde, vers saint Rémy, vers sainte Jeanne d'Arc et même vers Charles Martel

ou non, au chevet de Notre-Dame de Paris martyrisée, tout nous rappelle que la France reste la fille aînée de l'Église et que ce sont la sagesse de cette Église et le bras ferme de l'État qui permettent, encore aujourd'hui, à notre République de rendre « à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », comme l'a dit, le premier, voilà un peu plus de deux mille ans, un célèbre fils de charpentier

Pour empêcher le relativisme amnésique et le recul de la liberté des associations mixtes et diocésaines, il est nécessaire, juste et historiquement justifié d'adopter cet amendement. Quel est l'avis de

cet article n'a absolument pas pour objet de soumettre tous les cultes à une seule organisation, celle des associations cultuelles. Il ne remet pas non plus en cause les associations diocésaines spécifiques au culte catholique, qui résultent d'un accord international. le rappelle, cet article du projet de loi entend moderniser les règles de fonctionnement des associations cultuelles régies par la loi de 1905.

Le respect, la tolérance, la neutralité et l'impartialité sont des notions de premier plan qu'il nous faut utiliser pour élaborer une définition des associations à vocation cultuelle, vocation dont seul le préfet appréciera la qualité. Allons plus loin dans la clarification ; l'uniformité et l'application n'en seront que meilleures et la distinction avec les autres types d'associations, comme les associations mixtes, Soyons rigoureux dans nos termes : une association cultuelle ne doit viser que la célébration et l'accomplissement de cérémonies, rites et pratiques par des individus réunis dans la même croyance religieuse. L'amendement

La notion de culte, élaborée au regard des travaux parlementaires de la loi de 1905, est désormais parfaitement stabilisée dans la jurisprudence : il s'agit de la « célébration de cérémonies organisées en vue de l'accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de

et à l'entretien du culte. La définition proposée ne tiendrait en outre pas compte des associations diocésaines, dont nous avons parlé à propos de l'amendement précédent, qui ont justement la spécificité de ne pas avoir pour compétence d'exercer le culte. En effet,

personne n'a jamais non plus défini exactement ce qu'était un ministre du culte ; d'où la grande difficulté que nous avons avec nos compatriotes musulmans, car nous calquons sur l'imam la notion de ministre du culte que nous connaissons, celle des cultes précédents, alors que l'imam ne correspond pas au ministre des cultes tel que l'imaginent les chrétiens ou les juifs.

ni à l'esprit du législateur libéral de 1905. Au contraire, cela viendrait extrêmement contraindre la liberté de croyance et la liberté de culte dans notre pays, pour les cultes passés, les cultes présents, mais aussi, peut-être, pour les cultes à venir. Après tout, vous connaissez sans doute cette citation, on dit que « le christianisme est une secte juive qui a réussi ». Qui sommes-nous pour juger, d'un point de vue totalement laïque, de la réussite, de la vérité de la reconnaissance de tel ou tel culte ? Je pense que la République doit se garder d'avoir de telles opinions, même lorsque celles-ci sont fondées sur de bonnes intentions,

la qualité de votre argumentation, dont nous partageons totalement la première partie. Tout d'abord, la loi de 1905 a été réalisée par référence aux quatre cultes statutaires

Même si chacun peut avoir une opinion à cet égard, on sait que ce n'est pas à l'État d'expliquer s'il faut parler latin ou arabe dans les lieux de culte ! Cela pose des questions importantes, mais qui ne relèvent pas de la police administrative. La police des cultes désigne le fait que l'État ne reconnaît aucun culte, puisqu'il les reconnaît tous. Indépendamment du fait qu'il y a une qualité de culte et de liberté de réunion, il y a des avantages associatifs permis par la loi de la République. Ces derniers, qui sont importants, méritent, conformément aux principes que nous avons définis ensemble, notamment le non-subventionnement, d'entrer ou non dans tel ou tel critère. Si je puis me permettre, monsieur le sénateur, je pense que vous faites une légère confusion. Ce n'est pas parce que l'Union des athées ou les Témoins de Jéhovah réclamaient la possibilité d'être une association loi de 1905

que l'on bénéficie, sous le statut de 1905, des avantages réservés au culte, que n'ont pas les autres associations. Ainsi,

Tout aux croyants en tant que culte, mais rien aux croyants en tant que force politico-culturelle ». Tel est l'objet exact de notre texte. Je reconnais qu'il est original dans le concert des nations, mais c'est ce qui fait, je crois, la grandeur de notre pays.

Si nous sommes tous ici favorables au maintien de l'ordre public, il nous est pour autant difficile de comprendre en quoi celui-ci concerne les associations. Ce dispositif issu des travaux de la commission des lois et dont les modalités sont juridiquement floues et imprécises inquiète les représentants des cultes eux-mêmes. Prenons l'exemple d'une association cultuelle souhaitant venir en aide à une personne sans papiers au nom du devoir de fraternité. Pourrait-elle être considérée comme transgressant l'ordre public ? Est-ce la volonté de la Haute Assemblée ?

N'agissait-elle pas simplement, elle aussi, conformément au principe de fraternité, principe républicain par excellence ? Ce dispositif constitue une nouvelle fois un empiètement du politique sur le religieux. Il porte le risque d'un renforcement global du contrôle social auquel s'oppose le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires. Pour l'ensemble de ces raisons, nous en demandons la suppression. Quel est la commission ? Cet amendement vise à supprimer l'interdiction pour les associations cultuelles de troubler l'ordre public par leur objet statutaire ou par leurs activités effectives.

nous ont dit que ce genre de rédaction créait une sorte de suspicion. Il va de soi, monsieur le ministre, que l'ordre public doit être respecté ; ce n'est pas à vous que je vais le

monsieur le ministre.

J'ai déjà eu l'occasion de dire que la vraie mesure républicaine eût été sans doute, dans la philosophie de la loi de 1905, la nationalisation de tous les biens religieux, comme on l'a fait pour l'Église catholique à l'époque. Mais je pense que nationaliser les mosquées aurait été politiquement plus compliqué et, d'ailleurs, sans doute mal accepté par la majorité sénatoriale.

Le principe de non-subventionnement n'est donc pas un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Il se pourrait que le Conseil constitutionnel- je ne voudrais pas lui donner des idées, parce que, comme le dit la chanson, tout serait à recommencer pour le ministre de l'intérieur -considère que

je voudrais souligner que tout le monde a touché le chômage partiel dans les cultes, sauf les ministres du culte, quelle que soit la vie associative. Troisièmement, le principe de non-subventionnement est un principe législatif, mais non supralégislatif.

religieuses ». Il s'agit des « activités des organisations religieuses ou des particuliers fournissant des services directement aux fidèles dans les églises, mosquées, temples, les synagogues et vous nous dites que Bercy fait une différence, dans cette catégorie générale, entre les ministres du culte spécifiquement et ceux qui participeraient à l'exercice du culte et qui seraient laïques.

ayant notamment pour compétence de décider de l'adhésion de tout nouveau membre, de la modification des statuts, de la cession de tout bien immobilier

L'article 26 de ce texte prévoit, à son alinéa 5, que toute nouvelle adhésion d'un membre d'une association cultuelle doit être soumise à une décision d'un organe délibérant. En imposant ce fonctionnement aux associations, le présent article représente non seulement une véritable immixtion dans l'activité des cultes, mais aussi une contradiction au principe de liberté d'association. ainsi contraire au principe de la séparation de l'Église et de l'État. Il convient de laisser aux cultes la liberté d'organiser le choix des modalités de recrutement de leurs officiants. Ce dispositif est totalement disproportionné au regard de l'objectif apparent de cette loi, qui entend lutter contre le séparatisme lié à l'islamisme radical. Jusqu'où ira ce gouvernement ? Sera-t-il prêt à s'enfoncer dans cette obsession que représente désormais l'islam ? Et combien de principes aura-t-il reniés, pour ce faire ? Par conséquent, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires demande la suppression de cette disposition. L'amendement

que ces dernières seraient contraires à la liberté d'association. Or le Conseil d'État a rendu un avis précisant que ces dispositions tendaient à protéger la liberté de conscience et ne portaient pas une atteinte disproportionnée aux libertés de culte et d'association. Je rappelle que ces dispositions obéissent à un objectif d'intérêt général : protéger les associations contre d'éventuelles prises de contrôle par une minorité et assurer une meilleure information de leurs membres sur la gestion de leur patrimoine immobilier et sur le recrutement de leurs officiants. La commission

l'idéologie ... Ces trois principes, vous les connaissez. Premièrement, la liberté du culte est intégrale. D'ailleurs, elle est garantie par l'État et par la laïcité. Deuxièmement, il ne revient pas à l'État d'organiser les cultes. pourquoi nous demandons la suppression de cet alinéa. La loi n'a pas pour mission d'organiser les cultes. Ceux-ci s'organisent librement. Troisièmement, l'État veille à l'application de la loi, y compris dans la sphère religieuse. S'il y a des violences, s'il y a des coups d'État dans les religions, s'il y a des atteintes à l'ordre public, l'État doit intervenir.

conformément d'ailleurs à ce qui nous a été dit par nombre de représentants des cultes durant les auditions, de supprimer tout ce qui a trait à l'organisation des cultes. En revanche, nous sommes tout à fait scrupuleux sur ce point : la liberté, y compris celle de pratiquer ou de ne pas pratiquer un culte, doit être affirmée, et l'État en est le garant.

le culte. Là, vous infantilisez les religions, vous intervenez dans la vie des associations cultuelles et vous vous éloignez de la loi de 1905 vous représentez un État faible, et vous voulez entrer dans les méandres des associations pour donner le la ; soit la République est forte, responsable, et elle laisse le culte s'organiser ! Voilà ce que j'avais à vous dire.

Mme Esther Benbassa. Le présent article transforme la procédure actuelle de rescrit administratif en une obligation de déclaration auprès du préfet de la qualité cultuelle des associations Si la commission des lois a tenté d'améliorer le dispositif, en introduisant plus de souplesse lors du renouvellement des demandes des associations dont la qualité cultuelle aura déjà été reconnue pour une première période de cinq ans, et cela en prévoyant une simple obligation d'information de l'administration au bout de ces cinq années, il reste qu'une telle mesure se fonde sur une suspicion injustifiée et généralisée à l'égard des associations cultuelles. Il n'appartient pas à l'État d'organiser les cultes et d'opérer un contrôle permanent sur ceux-ci. L'article 27 a pour effet d'alourdir les contraintes administratives des associations cultuelles. C'est aussi une manière d'entraver la liberté des cultes, des cultes, qui n'ont pas toujours les moyens administratifs d'effectuer de telles démarches. En outre, ce contrôle renforcé est contraire aux principes qui découlent de notre laïcité, et il constitue un dévoiement de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l'État. Pour toutes ces raisons, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires en demande la suppression. Quel

C'est une rupture par rapport au système de la loi de 1905. Notre amendement a pour objet de rester dans un régime de déclaration unique, conformément à la loi de 1905, que nous connaissons un peu, monsieur le ministre, même si nous raisonnons par rapport à la France de 2021

qu'elle souhaite continuer à bénéficier de la reconnaissance de sa qualité cultuelle. La logique de la loi de 1905 est que cela figure dans les statuts.

Au-delà du lourd formalisme que cela représente, ce nouveau dispositif ferait apparaître une nouvelle catégorie d'associations de la loi de 1905 ne bénéficiant pas des avantages propres aux associations cultuelles- avantages dont les contours paraissent flous en l'état actuel du texte. » La Commission nationale consultative des droits de l'homme a aussi noté cette grande difficulté : « Serait ainsi créée, à côté des associations à objet cultuel de la loi de 1901 et de la loi de 1905, une troisième catégorie, celle des associations de la loi de 1905 ne bénéficiant pas des avantages propres à ce cadre législatif, dont le régime juridique reste à préciser. J'ajoute que la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour avoir violé l'article 9, alinéa 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, en appliquant à des groupes sectaires des dispositions fiscales dont la portée était insuffisamment précise. Monsieur le ministre, chers collègues,

proposons d'alléger la procédure, qui serait très contraignante avec ce renouvellement, en excluant les associations cultuelles déclarées avant l'entrée en vigueur de la Certes, l'article 45 du projet de loi prévoit une entrée en vigueur progressive, mais cela ne concernera en réalité qu'une partie des associations ayant acquis

au bénéfice des avantages découlant de la qualité d'associations cultuelles s'il constate que l'association n'entre pas dans cette catégorie.

monde associatif : « Cette procédure sera moins contraignante pour les associations tout en permettant à l'administration d'atteindre le même objectif en se consacrant à l'examen des cas les plus litigieux.

distinguer réellement ce qui relève du cultuel et qui doit être aidé et ce qui relève du culturel et qui n'a rien de religieux.

tacite de la déclaration initiale de qualité cultuelle d'une association auprès du préfet, que celui-ci pourrait écarter selon son bon vouloir. Il constitue une nouvelle attaque contre la liberté de culte et vient compliquer une procédure préexistante, puisque les associations culturelles sont déjà soumises à une obligation de déclaration préfectorale. Le présent amendement de repli a donc pour effet d'alléger la procédure, en demandant une reconduction tacite et sans condition de la reconnaissance de la qualité culturelle d'une association pour une durée de cinq années supplémentaires. Le renouvellement de la déclaration de la qualité culturelle d'une association se produira ainsi tous les dix ans. C'est le délai que nous proposons à l'alinéa 5 constitue une nouvelle fois un empiètement du politique sur le religieux, une atteinte au principe de séparation des Églises et de l'État. Le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires en demande donc la suppression. L'amendement

Après quinze ans d'existence, la qualité cultuelle fait l'objet d'une reconduction tacite à chaque échéance de cinq ans, sauf si, deux mois, auparavant, le représentant de l'État dans le département invite l'association concernée à renouveler la procédure de déclaration dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article. Il s'agit d'un compromis, mais qui a tout de même pour objet de simplifier le dispositif.

donc un avis défavorable sur cet amendement. L'amendement n° 449 rectifié a pour objet d'exempter du nouveau régime de déclaration les associations cultuelles déjà constituées avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Nous sommes pour le renouvellement

La procédure prévue par le projet s'apparente donc à une barrière à l'entrée du statut d'association cultuelle. Un tel régime porte une atteinte certaine au régime actuel, en vertu duquel les associations, y compris cultuelles, se constituent librement. » On sent qu'il y a là une interpellation du Conseil constitutionnel. Le président Retailleau, à propos de l'instruction en famille, nous a dit : « Un régime

Ce qui m'inquiète dans cet article, c'est que vous jetez une suspicion de principe sur l'exercice du culte. Je crains que cela n'entraîne, dans une partie de la population, un rejet massif

que la rédaction initiale. Il y a bien, non pas une autorisation, mais un contrôle du préfet. C'est déjà une meilleure base et un signe de moindre défiance. Je comprends l'objectif et la problématique du rescrit fiscal. Cependant, je comprends moins, monsieur le ministre, que l'amendement du Gouvernement vise à supprimer l'alinéa 5, qui a été rédigé par la commission des lois du Sénat.

même envoyer un courrier, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment une tacite reconduction, dans la mesure où elle doit malgré tout se signaler. Une fois qu'elle s'est signalée, le préfet, qui, effectivement, a pu changer, éventuellement, même, à la demande des élus, et qui découvrirait ces associations,

et à assouplir légèrement l'octroi des garanties d'emprunt, désormais possible sur toutes les communes du territoire, et non plus seulement dans les agglomérations en développement. Nous sommes favorables à cette disposition, car elle permettra un meilleur contrôle des constructions des nouveaux lieux de culte par les fidèles et par les pouvoirs publics. L'assouplissement de certains financements par garantie d'emprunt semble également bienvenu. Une telle mesure était réclamée par certains représentants des cultes reçus en audition,

de vérifier la qualité cultuelle de l'association, au moyen de la déclaration préalable qui lui est imposée pour bénéficier des avantages que sont la possibilité de contracter des baux emphytéotiques ou le bénéfice d'emprunts garantis par les communes, départements, etc. Je ne vais pas répéter ce que vous avez très bien dit vous avez défendu votre position. En outre, cette qualité est attribuée pour une durée de cinq ans, et l'article 27, tel qu'il a été voté à l'instant, assure un droit de suite de ce contrôle, car, avant le terme de cette échéance, l'association qui souhaite continuer à bénéficier des effets de la qualité cultuelle doit en informer le préfet deux mois avant l'expiration

Il ne vous est pas interdit de faire de la politique, mais, tant qu'à faire, autant que ce soit nous qui le rappelions, puisque vous avez oublié de le dire. La parole est à M. le ministre.

disons les choses très clairement : les élus communistes à la mairie de Strasbourg ont voté contre cette subvention à l'association Millî Görüs, parce que nous considérons qu'elle est le faux-nez en France du gouvernement Erdogan, qui vise l'implantation d'une politique néo-ottomane, nationaliste

à une association très peu recommandable, à savoir l'Union des musulmans de Rouen, affiliée aux Frères musulmans, qui tenait un séminaire pour les parents et les enfants, avec un orateur tout à fait ciblé par vos services. Lorsque j'en ai été informée, j'ai tout d'abord prévenu le préfet, lequel n'était pas au courant, puis j'ai saisi la mairie, qui, apparemment, n'était pas non plus au courant, mais qui avait tout de même accordé une salle. Plus on prévoira d'informations préalables, plus on mettra de contraintes,

avec les services de l'État par le passé. Elle a obtenu des contrats et des subventions, comme l'a indiqué la préfecture du Bas-Rhin. Cela a été confirmé par le journal. En mai 2020, la préfecture lui a accordé une subvention de 2 500 euros 2 500 euros au titre de la solidarité aux actions associatives lors du premier confinement. Par ailleurs, dans le cadre d'un partenariat institutionnel, une convention pour lutter contre l'insécurité routière dans les quartiers prioritaires strasbourgeois a été signée en 2020 entre cette association et

aux musulmans d'origine turcophone de Strasbourg et de son agglomération de disposer d'un lieu de culte satisfaisant. Il est quand même curieux, vous en conviendrez, qu'il n'y

financer par un bail emphytéotique ou une garantie d'emprunt l'extension d'un lieu de culte. Monsieur le ministre, vous nous proposez donc d'étendre à tout le territoire national une pratique qui est aujourd'hui réservée aux agglomérations dites en voie de développement.

Sylvie Vermeillet. La législation en vigueur autorise les collectivités territoriales à conclure des baux emphytéotiques avec les associations cultuelles pour la construction d'édifices cultuels. Le recours à cet outil est assez répandu parmi les communes, notamment dans les territoires caractérisés par un coût élevé du foncier.

À l'échéance du bail emphytéotique, l'édifice revient dans le patrimoine de la commune, ce qui peut constituer une contrainte pour celle-ci en raison des charges d'entretien et, parfois, de réparation du bâtiment

estimé que cet outil pourrait de la sorte représenter une bombe à retardement pour les collectivités concernées. C'est pourquoi M. Maurey préconise, dans ce rapport, de faciliter la cession de l'édifice aux associations cultuelles à l'issue du bail,

de la loi de 1905, les collectivités publiques ne peuvent pas financer la construction ou l'aménagement d'édifices cultuels. Cependant, l'article L. 1311-2

et donne au locataire les prérogatives du propriétaire durant la durée du bail. Dans un tel cadre, le prix payé est souvent modique : à l'expiration du bail, l'édifice construit revient à la collectivité publique. Il est donc parfaitement assumé que de tels contrats constituent une forme de subventionnement de la construction d'un édifice cultuel, en dérogation à la loi de 1905. Il s'agit cependant d'un outil bien identifié par le Conseil d'État, qui veille scrupuleusement à son application et appelle le plus souvent les parties à régulariser leur situation lorsqu'il constate des irrégularités dans les termes du contrat de bail. En outre, ce dispositif est efficace, surtout dans certaines parties du territoire où le coût du foncier est élevé : il a permis la construction de nombreux lieux de culte de toutes confessions. Toutefois, le régime légal en vigueur n'est pas sans inconvénient, dès lors que les collectivités ayant eu recours à un BEA redeviennent propriétaires du bâtiment à l'échéance du bail et qu'elles doivent alors de nouveau en supporter la charge, ce qu'elles ne souhaitent pas si leurs moyens sont limités. De son côté, l'association cultuelle perd alors l'usage de l'édifice cultuel. Dans le but de faire évoluer le cadre légal en vigueur, nous proposons donc d'inclure dans le contrat de BEA une option d'achat de l'édifice par l'association cultuelle à l'échéance du bail emphytéotique.

Nous comprenons en revanche que les collectivités territoriales préféreraient ne pas avoir autant de nouveaux lieux de culte à entretenir, puisque les églises dont elles sont aujourd'hui dépositaires sont déjà suffisamment lourdes à porter.

ce qui est tout à fait normal, à la suite de la plus grande nationalisation de l'histoire de notre République, celle qui résulte du décret du 2 novembre 1789 ! Voyez-vous, mes chers collègues, de temps en temps, même l'Église catholique profite des nationalisations révolutionnaires

Les conséquences juridiques, les analyses possibles, la façon même d'aborder cette problématique sont de fait très variées.

C'est pourquoi nous avons exprimé la position qui est la nôtre. La parole

du statut des associations. Nous défendons-là un amendement de suppression, car il nous semblerait de bonne politique de faire un bilan global

permet de se livrer à des activités commerciales et immobilières alors même que la loi de 1905 restreint strictement leur objet à l'exercice du culte. Il s'agit là d'une rupture de l'équilibre posé par l'article 19 de ce texte fondateur de la laïcité. la laïcité. Les nombreux avantages fiscaux dont bénéficient ces associations constituent des dérogations limitées au principe de séparation, liées à leur objet cultuel. Ces niches fiscales, qui font porter au contribuable une partie de la charge financière des cultes, ne sauraient être étendues à la gestion lucrative d'immeubles de rapport sans lien avec le culte.

dont la détention serait autorisée. Nous y voyons la reconnaissance par le Gouvernement du caractère anti-laïque de la mesure, dont il a tenté d'atténuer les effets, tout en le maintenant, malheureusement.

des associations relevant du domaine immobilier. Leur donner la possibilité de posséder et d'administrer des immeubles à titre gratuit, comme le prévoient les alinéas 5 et 6 de l'article

comment peut-on admettre que des associations cultuelles puissent tirer des revenus de la possession d'immeubles acquis à titre gratuit et qui ne seraient pas directement nécessaires à leur objet et à leur fonctionnement de base ? C'est une entorse à la loi originelle de 1905

Voudrait-on transformer peu à peu les organes bénévoles dédiés au culte en sociétés immobilières ?

et ajoute la possibilité pour les associations cultuelles de posséder et d'administrer des immeubles de rapport acquis à titre gratuit. Bien que cette disposition puisse être analysée comme un assouplissement notoire du financement des associations cultuelles, à compenser la baisse constante des dons des fidèles, elle ne nous paraît pas pertinente dans sa rédaction actuelle. En effet, il ne revient pas aux associations cultuelles d'administrer des biens immeubles acquis à titre gratuit. Ce n'est pas leur vocation que d'être des spécialistes du droit immobilier, de gérer des logements ou encore des locaux pour le compte d'autrui. En revanche, il est tout à fait légitime de considérer que des associations cultuelles ayant à leur disposition de tels biens, notamment par la voie de dons ou de legs, puissent en tirer des revenus qui seront par la suite dédiés à leur activité cultuelle. En plus de favoriser leurs ressources propres, cela remédierait à une différence de traitement existant de longue date entre les associations cultuelles et les associations d'intérêt public, tout en préservant leurs attributions respectives. En ce sens, cet amendement tend à ce que les associations cultuelles puissent désormais être libres de mettre à disposition des biens immeubles acquis à titre gratuit, ou d'en tirer un bénéfice foncier à destination de l'exercice

Cette restriction porte atteinte à leur liberté de gestion et risque de compromettre gravement l'équilibre financier de bon nombre d'entre elles. Le présent amendement vise donc à corriger cette inégalité de traitement et cette atteinte à la liberté,

du code général des impôts. Pour l'heure, sont imposables tous types de locaux meublés dédiés à l'habitation, à l'occupation à titre privatif de sociétés publiques ou d'organismes associatifs ou privés, ou à l'occupation d'organismes déconcentrés de collectivités territoriales. Les immeubles de rapport entrent pleinement dans ces cases. Sont-ils souvent des bâtiments servant aux exploitants agricoles ? Non ! Sont-ils souvent dédiés aux écoliers de pensionnat ? Pas trop ! Sont-ils souvent des résidences universitaires ? Un peu plus ... C'est pourquoi il paraît juste et normal que les propriétaires d'immeubles de rapport ne puissent être exonérés ni de la taxe foncière ni de la taxe d'habitation. L'amendement

alinéa 5, permet aux associations cultuelles de posséder et d'administrer des immeubles acquis à titre gratuit. Or les biens immobiliers des associations cultuelles sont aujourd'hui exemptés de la fiscalité afférente, notamment de la taxe foncière, ce qui s'apparente déjà à une forme de subventionnement déguisé, bien que cela soit justifié, en l'état actuel des textes, par l'objet social étroitement défini. Cette exemption se fonde sur le fait que ces associations ont pour objet exclusif l'exercice du culte. Il est donc indispensable que ce régime d'exemption ne soit pas étendu aux immeubles gérés en dehors de cet objet, sans quoi l'esprit de la loi de 1905 s'en trouverait violé. Le Gouvernement justifie son projet par

Si l'objectif d'assurer des ressources autonomes régulières aux associations cultuelles est légitime, ces dernières ne sauraient échapper au droit commun. Afin de répondre à cette attente, un amendement tendant à plafonner à 33 % la part des revenus locatifs que les associations cultuelles pourront générer dans le total de leurs ressources. Il a par ailleurs été précisé que les revenus locatifs des associations cultuelles seront assujettis à l'impôt, comme toute organisation qui possède des immeubles. Dès lors, il nous paraît nécessaire de compléter ce dispositif dans deux directions : d'une part, en inscrivant expressément dans la loi que ces immeubles non consacrés à l'exercice du culte sont bien soumis au droit commun fiscal

L'amendement n° 140 rectifié tend à exclure les immeubles de rapport du bénéfice des exonérations fiscales de taxe foncière et de taxe d'habitation.

Nous souhaitons conserver ce principe de non-subventionnement par l'État et les collectivités locales. Le second rail, celui que nous imposons et qui, à mon avis, marque une avancée très importante

55 % des Français ne payent pas d'impôt sur le revenu et nous savons tous que, quelles que soient les religions, les fidèles sont en moyenne plus pauvres que les autres. Souvent, les reçus fiscaux

indépendamment de l'argent venant de l'étranger, à la construction de l'Église ou du culte en question par des immeubles dits de rapport. Pour le coup, ceux-ci portent mal leur nom, puisque, par définition, ils ne rapportent pas grand-chose, si ce n'est qu'il s'agit d'un don gratuit.

également être prudentes : il faut empêcher toute possibilité d'accointances entre élus locaux et responsables d'associations vouées au culte. Si le droit de préemption est une prérogative de la collectivité territoriale, il ne serait pas acceptable que ce droit soit utilisé pour l'achat d'un bien ou d'un terrain qui serait par la suite revendu à une association cultuelle à un prix moindre, inférieur à celui du marché.

fins. Quel est l'avis de la commission ? La nécessité d'un tel amendement ne nous apparaît pas clairement. En effet, l'exercice par une personne publique de son droit de préemption doit déjà répondre à des objectifs d'aménagement ou d'urbanisme

du droit de préemption que vous évoquez, ma chère collègue, serait selon toute vraisemblance déjà illégal et la délibération procédant à une cession à vil prix en faveur d'une association cultuelle pourrait déjà être sanctionnée et déférée devant le tribunal administratif

permettrait une meilleure égalité cultuelle, tant du point de vue des obligations que des droits dont peuvent notamment bénéficier les ministres du culte des autres religions. Il est donc nécessaire que la question ne soit pas éludée et fasse l'objet d'un travail de fond dans les années à venir, en vue de régler ce traitement différencié des cultes.

de la plupart des contraintes administratives et comptables imposées aux associations relevant de la loi de 1905 et aux associations de droit commun loi 1901 qui ont une activité en relation avec l'exercice public d'un culte. public d'un culte. Selon l'étude d'impact, il s'agit d'inciter les acteurs du culte à s'organiser sous le régime des associations cultuelles et à séparer ainsi leurs activités cultuelles des autres. Malgré les efforts de la commission des lois, qui a souhaité exclure de ce régime d'obligations renforcées les associations 1901 dans lesquelles l'activité cultuelle n'a qu'un caractère strictement accessoire, celles-ci seraient désormais soumises au contrôle de l'administration. Les associations loi 1901, par exemple les organismes de gestion de l'enseignement catholique ou les mouvements de scouts, organisent des actes en relation avec l'exercice public d'un culte. Elles pourraient ainsi entrer dans le champ d'application de l'article 30 et se voir imposer des obligations très contraignantes. En outre, les nombreuses associations loi 1901 sont inspirées par des convictions spirituelles actions humanitaires, collectes alimentaires, aide aux personnes précaires ... Comment feront-elles, lors de leurs opérations comptables, pour faire le départ entre leurs activités en relation avec l'exercice public d'un culte et celles qui n'en sont pas ? Parce que ces mesures sont sans lien avec les réalités et les pratiques de l'exercice du culte en France, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires demande la suppression de cet article. Quel

le projet de loi prévoit que les comptes puissent être séparés et que la partie cultuelle soit soumise aux obligations de la

du champ d'intervention du ministère de l'intérieur les associations qui se déclarent culturelles, mais qui pratiquent des activités cultuelles. Les scouts disent qu'ils sont strictement accessoirement cultuels. Par exemple, l'Association interculturelle du Grand Nancy se présente dans son statut comme une association qui mène des activités culturelles, sociales, éducatives et sportives au sein de la communauté turque et française,

l'expose clairement : les associations gestionnaires des mosquées doivent être sous le régime de 1905. Il convient le cas échéant de séparer les activités cultuelles des activités

et un objet non cultuel. Si leur classification est différente, il y a cependant entre ces deux divisions d'associations de très nombreux points de convergence. Cet amendement vise donc à mieux encadrer les ressources financières des associations mixtes.

faire apparaître séparément la comptabilité relative à leurs activités cultuelles. L'amendement de notre collègue Delattre tend à proposer une amélioration rédactionnelle de cet article

l'avis du Gouvernement ? Nous sommes défavorables à l'amendement de Mme Delattre.

: La parole est à Mme Sylvie Vermeillet. Cet amendement d'Hervé Maurey a pour objet de compléter les mesures de transparence financière prévues par le présent article en soumettant tout projet de construction d'un édifice du culte par une association à objet mixte

fait au nom de la délégation aux collectivités territoriales en 2015, a pour finalité d'accroître la traçabilité des flux financiers à l'origine des projets d'édifices du culte. L'amendement tend à fixer les mêmes sanctions qu'en cas de non-publication d'un compte annuel par les associations cultuelles et les associations à objet mixte prévues par le présent projet de loi.

Merci,

: La parole est à M. Jean-Yves Leconte. L'article 30 du projet de loi a pour objectif de soumettre les associations mixtes, c'est-à-dire les associations de droit commun ayant un objet en partie cultuel, aux prescriptions d'ores et déjà applicables aux associations cultuelles telles qu'elles sont renforcées par ce projet de loi. L'échange que le ministre et la rapporteure ont eu sur l'amendement n° 652 du Gouvernement montre la complexité du sujet. Or, en l'état, cette disposition ne met en oeuvre aucune modalité permettant aux associations visées d'exercer leur droit à un recours juridictionnel. Cela est d'autant plus contestable qu'est ici en jeu l'effectivité de la liberté d'association, droit fondamental tant au titre du bloc de constitutionnalité que de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme Pour remédier à cette insuffisance, nous proposons d'ouvrir au bénéfice des associations cultuelles un recours en référé contre l'astreinte qui leur est adressée lorsque le préfet juge qu'elles n'ont pas satisfait aux exigences imposées. Il s'agit d'octroyer aux associations concernées une contrepartie aux très nombreuses exigences et obligations nouvelles qui s'imposeront à elles à l'entrée en vigueur de ce texte. Quel

sur le point de savoir à quel juge confier éventuellement cette mission. Ses cosignataires sont soucieux de préserver la liberté d'association et la liberté d'exercice des cultes

en référé, le pouvoir d'enjoindre sous astreinte à une association de mettre en conformité son objet avec la réalité de ses activités, en l'occurrence cultuelles.

de contrôle des associations et des subventions prévus aux articles L. 12 et L. 14 du livre des procédures fiscales. Évidemment, notre livre de chevet est le jaune budgétaire sur l'effort financier de l'État en faveur des associations :

qui nous permettra d'avoir une meilleure visibilité de l'ensemble des financements publics accordés aux associations.

nous semble collectivement important d'évaluer exactement et en toute transparence les modalités, les formes et les volumes des ingérences étrangères dans l'organisation des cultes

a reconnu le génocide des Arméniens. Il est insupportable qu'une association, quelle qu'elle soit, dont on comprend bien qu'elle est le faux-nez du gouvernement Erdogan, continue à perpétrer des actes contre la communauté arménienne.

dernier prévoit ainsi une astreinte pour les dirigeants de ces associations qui ne souhaitent pas produire leurs comptes annuels. Ces nouvelles contraintes nuisent gravement à la vitalité des petites et moyennes associations cultuelles. Enfin, il est curieux de penser que cette mesure sera utile pour lutter contre l'islam radical, objectif apparent de ce projet de loi. Dans la pratique, ce dispositif requiert une obligation de certification des comptes de la part des associations cultuelles. Or une telle opération est très lourde pour les petites associations. Les organisations confessionnelles parfaitement respectueuses des valeurs de la République seront ainsi soumises à de multiples complications bureaucratiques.

que la liberté de culte doit être intégrale, garantie par l'État et par le principe de laïcité. Il faut dire, redire et redire encore qu'il ne revient pas à l'État d'organiser les cultes,

la suppression de l'article 33, qui va alourdir considérablement la tâche d'un certain nombre d'associations.

-soit mentionné dans l'annexe des comptes annuels, sans toutefois y figurer. Le traité d'apport est bien souvent un document très volumineux : l'annexer risquerait à coup sûr de complexifier la lecture des comptes annuels

injuste, nous avons essayé d'obtenir des commissaires aux comptes des missions spécifiques. Nous proposons, par cet amendement, de fixer des seuils

Cet amendement vise à compléter les mesures de transparence financière prévues par le présent article en soumettant tout projet de construction d'un édifice du culte par une association cultuelle à l'élaboration d'un plan de financement prévisionnel, certifié par un commissaire aux comptes. dispositions de l'amendement n° 382 rectifié que nous avons adopté à l'article 30. Cette mesure viendrait utilement compléter les obligations de transparence qui pèsent sur ces associations en permettant de connaître, avec fiabilité,